citoyen et écologiste, de la proposition de résolution proposant au Gouvernement de sortir le système électrique des mécanismes concurrentiels, présentée, en application de l'article 34-1 de la Constitution, par MM. Fabien Gay, Pierre Laurent, Mme Marie-Noëlle Lienemann et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 176). Dans la discussion générale, la parole est M. Fabien Gay, auteur de la proposition de résolution. Monsieur

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, jour après jour, l'impact des prix de l'énergie sur les usagers, nos entreprises, nos collectivités territoriales donne à voir l'ampleur de la crise qui est devant nous. Le mythe de la libéralisation du secteur de l'énergie et de ses mécanismes concurrentiels, qui devaient faire baisser les prix, n'a pas passé l'épreuve de la réalité.

du marché européen de l'énergie et de ce mécanisme de construction des prix, de prendre un autre chemin que celui de l'Europe du marché et des. Nous voulons construire ensemble une Europe de l'énergie

Tout comme nous pouvons faire du commerce sans traités de libre-échange climaticides, puisque l'on commerce depuis l'Antiquité, nous pouvons maintenir les interconnexions et les échanges solidaires sans laisser les faire du profit. Mes chers collègues, le marché européen actuel ne peut pas fonctionner, car il repose sur trois illusions. La première est que l'électricité est une marchandise comme une autre et que l'on pourrait organiser de toutes pièces un marché où l'offre rencontrerait la demande. Sauf qu'un marché s'organise, certes, avec une offre et une demande, mais surtout avec un stock ! Si l'offre est supérieure à la demande, le prix est faible ; et inversement.

le système favorise le. Nous continuerons donc à dire que l'électricité, et plus largement l'énergie, parce qu'elles sont nécessaires à la vie, doivent être sorties du secteur marchand et reconnues comme un bien commun de l'humanité. J'aimerais ensuite revenir sur une deuxième illusion

ou à investir dans les énergies renouvelables. Car, quoi qu'il arrive, et même sans investissement, ils payeront le même prix que leurs voisins. Troisième illusion : le marché européen mettrait en lien producteurs et acheteurs. Mais là où il y a un marché,

Il faut arrêter ce massacre et ce racket organisé ! Oui, il est possible de faire autrement ! D'ailleurs, beaucoup de monde, même à droite, est désormais d'accord avec nous pour délier les prix du gaz et de l'électricité. Très bien ! Mais comment faire sans sortir de ce système ?

l'ensemble des consommateurs et des consommatrices et qui, surtout, repose sur un mix électrique national. Nous devons faire valoir notre intérêt, celui du nucléaire, mais nous devons aussi

madame la ministre, mes chers collègues, depuis près d'un an, le marché de l'énergie connaît des perturbations historiques, notamment en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022. Ce contexte international, inédit au XXIsiècle, place le marché énergétique en tension et a été le révélateur d'une crise du marché électrique sous-jacente. En effet, avec le système actuel, le avec le système actuel, le prix du mégawattheure a atteint des niveaux sans précédent, passant de 40 euros début 2021 à 400 euros en septembre 2022. De telles hausses, même si le prix du mégawattheure a eu tendance à baisser récemment, aux alentours de 137 euros, ne sont acceptables et supportables ni pour nos entreprises ni pour l'ensemble des particuliers. Elles s'expliquent en partie par le fonctionnement actuel du marché électrique européen, qui nous place en économie de guerre. En effet, le prix de l'électricité étant indexé sur celui du gaz, peu importe le coût réel de la production, le prix final dépend du contexte international que nous ne pouvons pas contrôler. S'il convient de noter les interventions de l'État pour contenir la hausse du prix de l'électricité à l'aide du bouclier tarifaire, du dispositif « amortisseur électricité » ou encore des chèques énergie, le problème de fond n'est pas réglé.

nous conduit aujourd'hui à vendre notre production électrique nucléaire à bas coût pour la racheter ensuite plus cher sur le marché européen. Ce système en pleine crise est une aberration qui profite aux revendeurs : ce sont les consommateurs français qui en payent le prix fort C'est d'autant plus vrai qu'il s'accompagne d'une extension progressive des tarifs réglementés de vente dont le coût se répercute, une fois de plus, sur nos concitoyens et sur les entreprises nationales. Rappelons d'ailleurs que les énergies renouvelables sont prioritaires lors de l'injection sur le réseau, ce qui conduit à presque arrêter les structures de production électrique pilotables lorsqu'il y a du vent notamment. Quelque part, cela nous fait payer deux fois la production, puisque nous n'avons pas la maîtrise du stockage de l'énergie. À l'inverse, lorsque les énergies renouvelables sont à l'arrêt, nous n'avons plus suffisamment de pilotable disponible à fournir, notamment à cause de l'Arenh, et nous payons jusqu'à dix fois le prix, ce qui est insensé À cela s'ajoute la mauvaise gestion interne d'EDF, avec un déficit financier structurel étalé sur plusieurs années. Cette situation particulièrement préoccupante contraint aujourd'hui l'État à reprendre la main. C'est aussi la gestion de l'entretien du parc nucléaire par l'entreprise qui nous place dans une situation complexe. Fin octobre, plus de la moitié du parc nucléaire était hors d'usage. En cause, des problèmes d'érosion sur des réacteurs qui ont nécessité une intervention rapide et fait émerger des critiques sur une potentielle négligence eu égard à l'entretien des centrales.

L'électricité n'est pas un produit de consommation comme un autre, elle ne doit pas dépendre uniquement de l'offre et de la demande. Tant pour sa production que pour sa disponibilité auprès des usagers, il importe de définir un cadre souverain devant dépasser les seules lois du marché. de résolution soumise à notre examen aujourd'hui vise à sortir le système électrique des mécanismes concurrentiels. S'il est une certitude, c'est effectivement que nous ne pouvons pas nous contenter du actuel.

: sans elles, ce sont des territoires, des services et une certaine qualité de vie qui sont menacés ! Il s'agit d'une préoccupation majeure dans chaque commune. Les maires doivent désormais choisir entre chauffer convenablement leur école, permettre à leurs administrés de faire du sport ou défendre des projets pour leur commune. Certains m'opposeront qu'au nom de la libre concurrence, nous ne pouvons plus aider nos collectivités financièrement. Soit. Mais nous devons nous battre collectivement pour leur permettre d'accéder à un tarif attractif ne faisant pas l'objet de spéculation, afin qu'elles puissent continuer d'exercer, pour ceux qui l'auraient oublié, leurs missions de service public parce que le monde économique est menacé. Réalisme ou défaitisme, le spectre d'un mur des faillites causé par la hausse des prix de l'énergie se dresse d'ores et déjà devant nous. Nos boulangers baissent le rideau, nos restaurateurs commencent à manifester leurs craintes, nos artisans arrivent à bout de leurs capacités, certaines grandes entreprises préfèrent ne plus produire et recourir au chômage partiel. Le marché européen nous asphyxie ! Je le dis clairement, si nous ne pouvons pas aider plus nos collectivités, nos particuliers, nos TPE-PME, c'est à la base du problème et avec courage qu'il faut s'attaquer ! Les Français nous le demandent Pour agir concrètement désormais, deux voies s'offrent à nous : une réforme du marché de l'électricité européen ou une sortie du marché européen, afin de contrôler directement les prix de l'électricité. Pour bien mesurer l'action à mettre en oeuvre, le premier point crucial est de s'interroger sur la place du nucléaire en France. Aujourd'hui, nous sommes pénalisés si nous n'utilisons pas assez d'énergies renouvelables alors même que l'électricité produite par la France est quatre fois plus décarbonée que celle qui est produite par l'Allemagne. Des pistes européennes existent, avec notamment une refonte du marché de l'électricité. Elles devront s'accompagner d'une réflexion approfondie sur la place que doivent prendre les différentes énergies, notamment les renouvelables et Une révision complète des règles relatives au marché européen de l'électricité a été annoncée par la Commission européenne le 18 octobre 2022. C'est une annonce salvatrice, mais qui tarde à être concrétisée dans les faits. Parmi les pistes évoquées ou actées lors des derniers conseils européens, on propose de découpler les prix du gaz et de l'électricité, afin de mettre fin au système du, qui conduit à une hausse artificielle du prix de l'électricité. également de plafonner le prix du gaz, et donc par extension de l'électricité, la bourse TTF, le marché gazier de référence à l'échelle européenne, mais le contexte international ne nous y aide pas. Au-delà, il y a également la piste pour la France de sortir temporairement du marché électrique européen. C'est une piste pertinente qu'il ne faut pas exclure. La dérogation temporaire aux règles du marché de l'électricité accordée aux deux pays de la péninsule ibérique peut faire des émules. Il convient malgré tout de noter qu'il s'agit d'une dérogation, donc une mesure d'exception, qui a été accordée eu égard au faible nombre d'interconnexions électriques du Portugal et de l'Espagne. La majorité du groupe Union Centriste estime qu'une sortie dérogatoire et temporaire du marché européen de l'électricité peut être opportune. Rien ne semble expliquer qu'un pays comme la France ne puisse en bénéficier également. Les mêmes opportunités doivent pouvoir être offertes à l'ensemble des États membres de l'Union

une résolution est l'outil parlementaire adéquat pour alerter sur le caractère européen de la problématique structurelle que constitue la crise de l'électricité. Nous avions également précisé que nous soutiendrions un texte sans idéologie ni dogmatisme qui mettrait en lumière les dysfonctionnements du marché européen de l'électricité. Si nous saluons la volonté et les objectifs initiaux des auteurs du texte, nous ne souscrivons aucunement à l'ensemble des propos tenus par les auteurs de cette proposition de résolution dans l'exposé des motifs. Un monopole et une économie administrée n'ont jamais permis de préserver durablement le pouvoir d'achat ... Nous ne prônons aucunement une fin de l'intégration européenne. Nous sommes en faveur d'un assouplissement des règles et d'une refonte complète de celles-ci. Tout cela est primordial.

Notre impréparation généralisée conduit à ce que les États soient dans l'obligation de répondre en urgence à des situations de pénurie. La prospective devient indispensable en matière de stratégie énergétique, qui doit pouvoir être souple tant les incertitudes sont nombreuses pour assurer notre sécurité d'approvisionnement, préserver nos concitoyens, maintenir la vie économique du pays et les emplois. Si l'électricité constitue un bien de première nécessité, comme l'a admis le Conseil d'État, ce statut n'a malheureusement pas été reconnu pour le gaz, justifiant ainsi en droit la suppression progressive des tarifs réglementés de vente. Les différents intervenants de la table ronde organisée au Sénat au mois de décembre dernier par la commission des affaires économiques l'ont souligné le marché européen a été conçu pour gérer l'abondance d'énergie. Depuis sa création, la situation a profondément évolué du fait d'une combinaison de crises sanitaire, géopolitique et climatique. Si les premières n'étaient pas prévisibles, la fin des énergies fossiles et le réchauffement climatique l'étaient bel et bien. Ainsi, le marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne peut pas être adapté à ces défis. Des économistes le reconnaissent, ce marché n'incite pas à l'investissement sur le long terme. Il ne répond plus aux promesses avancées au moment de sa création : meilleur coût pour les usagers, sécurité d'approvisionnement, indépendance énergétique.

L'intégration du coût d'approvisionnement des fournisseurs alternatifs sur les marchés de gros dans le calcul de ces tarifs pour assurer leur contestabilité provoque leur renchérissement.

Cependant, l'échec actuel du marché n'explique pas tout. Nous avons accumulé un retard considérable sur tous les fronts : renouvelable, nucléaire, efficacité énergétique, économies d'énergie ou résilience des réseaux. Que l'on préserve des mécanismes concurrentiels ou non, je ne crois pas, pour ma part, que les prix de l'énergie puissent artificiellement baisser. Ils doivent en effet couvrir les coûts de production, qui, eux, augmenteront dans les années à venir au regard du mur d'investissements qui nous attend. Il n'y a pas de magie ! Aussi, la sortie de la France du marché européen de l'énergie, plus qu'une solution, se révélerait fortement déstabilisatrice. Les échanges transfrontaliers doivent être maintenus, sinon développés. En attendant, assurons-nous que ces prix n'excèdent pas le coût de production auquel il serait ajouté une « marge raisonnable ». C'est le sens de l'adoption en loi de finances de la taxe sur la rente inframarginale, qui devrait rapporter entre 7 milliards d'euros et 11 Peut-on réellement conjurer la volatilité des prix et la spéculation ? Oui, je le pense. La piste des contrats de long terme pour d'autres énergies que les renouvelables semble avancer, afin de donner de la visibilité à tous les acteurs, de calmer le jeu et de permettre d'investir dans de nouvelles capacités de production avec un peu plus de sérénité. Certes, l'Union européenne n'a, pour l'instant, proposé que des solutions temporaires. Il est regrettable que chaque État membre continue de négocier des dérogations dans son coin, créant une concurrence faussée.

renouvelables. Le et la détermination du prix de l'électricité par le coût de la dernière centrale appelée, le plus souvent le gaz, leur bénéficie pleinement ! La réforme doit être étudiée et discutée, afin de dessiner un mécanisme à la fois juste et solidaire au niveau européen. Surtout, le Parlement devrait être informé de manière permanente de l'état de ces négociations et des solutions envisagées. Le Gouvernement plaide à l'échelon européen pour une décorrélation décorrélation du prix de l'électricité de celui du gaz, pour un plafonnement du prix de l'énergie sur le marché de gros, qui vient d'être acté, mais la réalité est surtout que la demande est supérieure à l'offre. Ce problème de volume ne constitue pas une situation provisoire. Aussi, la solution à la flambée des prix de l'énergie n'est pas aussi simple que de sortir le système électrique des mécanismes concurrentiels, ni techniquement, ni économiquement, ni juridiquement. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, délestage, blackout, sobriété, et même col roulé : depuis plusieurs mois, les Français sont bercés, pour ne pas dire inondés, d'un verbatim anxiogène. Cela fait craindre, dans l'immédiat, un passage difficile de l'hiver et des factures énergétiques qui explosent. Et cela interroge sur les raisons profondes d'une telle situation. Reconnaissons que personne ne prêtait vraiment attention aux comparatifs de coût de l'électricité, historiquement très favorables à notre pays, qui montraient régulièrement un rapport d'un à trois, par exemple, avec nos voisins allemands. Encore moins nombreux étaient ceux qui s'intéressaient de près à la raison de ce différentiel important pour la commercialisation des électrons si essentiels à notre vie de tous les jours. Il a fallu la violence d'une crise énergétique sans précédent, ou presque, pour comprendre le mécanisme infernal dans lequel la France s'est fourvoyée. Chacun a bien compris maintenant que l'électricité pouvait être produite par différents moyens : nucléaire, hydraulique, éolien, photovoltaïque, biomasse, gaz, pétrole et charbon. De l'option choisie dépendent le coût de la production et son impact environnemental, chaque pays faisant son choix en fonction de potentiels propres et de données géopolitiques parfois anciennes. C'est particulièrement vrai sur notre continent. Ainsi, l'Allemagne a hérité d'un approvisionnement en gaz russe, relativement bon marché, mais très émetteur de CO2, tout en s'appuyant sur des centrales à charbon au bilan écologique inversement proportionnel au rendement économique. De son côté, la France s'est orientée dès les années 1950 vers le nucléaire, très bon marché et très faiblement carboné, contribuant progressivement à assurer sa souveraineté dans le domaine. En quelque sorte, chacun avait choisi sa stratégie pour composer son mix électrique, sans solliciter une quelconque autorisation auprès de l'Union européenne, tout en s'associant

surprise ! Il n'est pas judicieux de remettre en cause le mécano énergétique que j'ai décrit. Ce marché unique de l'énergie est en plein accord avec les principes fondamentaux de la construction européenne. On peut On peut même admettre que cela constitue un certain équilibre dans un réseau ainsi interconnecté, du fait de logiques différentes dans la production faisant appel à des sources d'approvisionnement diversifiées. Mais c'est Mais c'est ailleurs que le bât blesse : marché unique ne signifie pas tarification unique ! À quel moment avons-nous accepté de fixer nos coûts de production sur ceux, nettement moins avantageux, de pays certes partenaires, mais qui doivent pouvoir assumer seuls leurs propres stratégies ? À quel moment a-t-on accepté de lier les destins électriques de pays aux orientations divergentes en se basant sur les moins vertueux ? S'il y a bien une chose que l'on n'attend pas de la construction européenne, c'est qu'elle mette à mal des stratégies industrielles nationales ou qu'elle sacrifie un avantage concurrentiel. C'est pourtant exactement ce qui a été scellé, certes de manière discrète, mais néanmoins sournoise, avec la tarification européenne de l'énergie. En indexant le coût de l'électricité sur celui du gaz, au motif qu'il s'agirait de la dernière énergie capable de produire notre électricité en cas de pénurie, on bafoue complètement notre souveraineté, savamment construite par le président Pompidou dans les années 1970. C'est un peu comme si le prix des agrumes était indexé sur le coût de production dans les pays baltes au seul motif qu'il s'agirait d'une main-d'oeuvre plus facilement mobilisable en dernier recours, sans considération particulière quant à la météo dans ces pays. C'est Ce mécanisme de calcul intègre le coût sur le marché de gros, soumis à de fortes fluctuations depuis l'automne 2021, et de manière encore plus aiguë depuis le conflit en Ukraine, dont l'une des conséquences est l'envolée du prix du gaz, liée à l'arrêt de l'approvisionnement russe. De surcroît, ce tarif calculé n'est absolument pas capé, d'où des cours instantanés totalement délirants jusqu'à 2 000 euros le mégawattheure ! Cette situation n'est d'ailleurs pas sans rappeler

Certes, soyez tranquilles, le président Macron a bien identifié le problème et promis de convaincre ses collègues européens de revenir sur ce mécanisme, à l'instar de l'Espagne et du Portugal, qui ont atteint cet objectif avec moins d'emphase, mais bien plus d'efficacité ... Pour quel résultat à ce jour ? Le communiqué du dernier Conseil européen est impressionnant : « Le mécanisme de correction du marché sera automatiquement activé si " l'événement de correction du marché

une vraie prouesse technocratique ! Il faut vraiment en finir avec cette tarification absurde qui piétine toute politique nationale, aussi judicieuse soit-elle. Imaginez un peu, mes chers collègues, si jamais nos dirigeants avaient continué sur la voie pompidolienne, nous serions non pas les rois du pétrole, mais les empereurs de l'électricité, et notre modèle énergétique s'imposerait vraisemblablement à l'ensemble du continent européen

Sans doute nostalgiques d'une économie totalement administrée, qui n'a pourtant pas, à travers l'histoire mondiale, rencontré le succès escompté, vous accablez le caractère libéral du marché européen. Mais, en vérité, c'est seulement le mécanisme de l'Arenh qui est en cause, à savoir livrer à des fournisseurs une partie de la production de l'opérateur historique au prix concurrentiel de l'électricité d'origine nucléaire, quasiment sans aucune contrepartie et sans aucun algorithme de réajustement en fonction de la conjoncture. La véritable ouverture à la concurrence consisterait à permettre à des producteurs de proposer leurs propres tarifs de fourniture, dans une logique d'optimisation des coûts complets, dont les bénéficiaires seraient en définitive les consommateurs. Nous sommes très loin de ce schéma, qui, d'ailleurs, ne vous conviendrait sans doute pas davantage.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la crise énergétique que nous traversons nous fragilise considérablement. Nos ménages sont fortement impactés, nos entreprises et tout le tissu entrepreneurial sont menacés. La compétitivité de notre pays et, plus largement, celle de l'Union européenne seront fortement affectées. Il est impératif que l'Union sorte de sa dépendance aux énergies fossiles, en provenance particulièrement de la Russie. À ce titre, le plan REPowerEU est un outil intéressant. Il repose sur un triptyque simple : faire en sorte d'effectuer des économies d'énergie, diversifier nos sources d'approvisionnement en énergie et, surtout, produire notre énergie de manière propre.

Un paquet vert se met en place au fur et à mesure depuis 2019, traduisant une volonté de transition écologique. La transition énergétique en fait partie. Des réponses arrivent également concernant la crise actuelle, malgré des difficultés visibles lors des conseils européens tout au long de l'année 2022. Le 22 décembre dernier, un règlement dit « d'urgence » établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables a été publié au. Le texte est d'application directe pour les dix-huit prochains mois. Le travail des États membres de concert avec l'Union européenne constitue une véritable valeur ajoutée. Le marché intérieur européen de l'énergie est une force, mais il n'est pas abouti, et la réforme structurelle annoncée est plus que nécessaire. Tout d'abord, parce que si les craintes sont fortes pour cet hiver,

importants pour la France, puisqu'il permet de ne pas manquer d'énergie et de revendre l'énergie que nous produisons. Cette année est particulière pour nos installations nucléaires, mais n'oublions pas, à l'heure où l'on travaille à leur relance, que nous revendons aussi beaucoup sur le marché européen de l'énergie. Je salue l'implication du Gouvernement sur le principe du découplage du prix du gaz et du prix de l'électricité. Notre groupe soutient ce découplage et l'appelle de ses voeux depuis plusieurs mois. De manière générale, nous soutenons la réforme du marché européen de l'énergie. Mais ce que notre groupe ne souhaite absolument pas, c'est une sortie de fait de ce marché : les difficultés seraient alors bien plus grandes

de stations de transfert d'énergie par pompage (Step). Hier matin, en audition devant la commission des affaires économiques, Mme la ministre a été transparente sur la volonté de stratégie avec le nouveau patron d'EDF pour aborder les négociations à venir avec la Commission européenne. L'hydroélectricité fait partie de notre avenir et de notre souveraineté. Elle est gage de notre indépendance énergétique. Cependant, pour toutes les raisons évoquées

Le vidéaste Heu?reka a tenté d'expliquer le marché commun européen de l'électricité, auquel, soyons francs, presque personne ne comprend rien, pas même le ministre de l'économie, qui oscille entre approximations et contre-vérités Là où une vidéo de vulgarisation dure généralement quelques dizaines de minutes, il a fallu à notre vidéaste quatre vidéos et plus de trois heures trente d'explications pour venir à bout du marché de l'électricité.

À l'époque, il était possible de croire que le mécanisme de libéralisation permettrait d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables (EnR), totalement délaissées par EDF, enfermé dans sa stratégie du tout nucléaire, dont les limites sautent chaque jour un peu plus aux yeux. ans plus tard, force est de constater que le compte n'y est pas. Le marché européen était censé offrir le meilleur prix au consommateur. Au lieu de cela, comme le prix est commun et comme les opérateurs refusent de faire tourner leurs centrales à perte, il instaure, de fait, un prix unique basé sur le coût de production de la dernière centrale mobilisée, le plus cher du continent. Le marché était censé favoriser la multiplication des producteurs-fournisseurs d'énergie, particulièrement en matière de renouvelable : il a essentiellement créé des fournisseurs qui ne produisent rien et se « gavent » sur le dos du contribuable grâce aux tarifs réglementés et à l'Arenh. Pour le développement de la production d'EnR notamment, les règles de marché étant structurellement inadaptées, l'État a eu recours à des contrats de long terme à prix garanti avec les opérateurs. D'une manière générale, ouvrir à la concurrence les monopoles naturels et multiplier les acteurs privés utilisant la même infrastructure publique unique est une curieuse idée dont on a vu toutes les limites avec le rail. Il faudra- hélas ! -encore quelques années à certains pour s'en apercevoir. Pour l'électricité, qu'il faut à chaque instant produire dans des quantités suffisantes, mais sans surplus, multiplier les acteurs privés avant tout soucieux de leurs marges sur un réseau interconnecté reliant une trentaine de pays relève tout simplement de l'inconscience. Résultat des courses : une spéculation débridée et des tarifs totalement déconnectés des coûts de production. C'est encore une fois l'État, à coups de bouclier tarifaire, qui vient amortir cette inconséquence. L'échec est complet à part quelques libéraux dogmatiques confinant au fanatisme, tout le monde le concède ! Malgré quelques réticences, les États membres ont enfin décidé de restructurer le marché unique de l'électricité. Mais ni la proposition de la Commission de plafonner à 200 euros par mégawattheure les prix d'achat aux producteurs disposant des centrales les moins chères ni la proposition française de développer des contrats à long terme publics ou privés ne semblent à ce de protéger les consommateurs de la volatilité des prix ou de sécuriser les investissements nécessaires à la transition énergétique. Ces propositions ne sont pas à la hauteur de l'attente des artisans,

Elles ne sont également pas à la hauteur de l'urgence de la transition énergétique, qui demande de la visibilité à moyen et long termes pour tous les acteurs. Seule la puissance publique est en mesure de réguler les prix payés par les consommateurs en harmonisant les coûts très variables d'un type de production à l'autre et de planifier les investissements nécessaires à la transition. L'énergie n'est pas une marchandise comme les autres ; c'est un bien commun dont la fourniture à prix régulé doit être garantie. C'est le sens de la proposition des écologistes lors de l'élection présidentielle de remettre à plat des directives européennes. Je précise au passage que contrairement à ce que veut bien raconter le ministre, suspendre ou sortir du marché commun de l'électricité, ce n'est certainement pas mettre un terme à la solidarité ou au commerce d'électricité entre pays européens, qui existait avant et existera après le marché unique. C'est le sens également de notre proposition de renationaliser EDF pour en faire le bras armé de la transition énergétique, de notre volonté de conserver les barrages hydroélectriques dans le giron public et de notre proposition de loi visant à créer un service public des énergies renouvelables. Le groupe écologiste partage les principaux objectifs de cette résolution. En rappelant son attachement viscéral au respect de la règle commune européenne, il demande au Gouvernement de plaider avec force à Bruxelles pour une remise à plat totale des mécanismes concurrentiels. Dans ces conditions, il apporte son soutien à cette proposition de résolution.

Au-delà des imperfections liées à la manière dont nous avons procédé, en France, à la libéralisation, pour nous conformer aux directives européennes ouvrant les secteurs de la production et de la fourniture d'électricité à la concurrence, rappelons concurrence, rappelons que, si les prix de l'énergie ont atteint des sommets en 2022, c'est essentiellement en raison de l'agression de l'Ukraine par la Russie et de l'utilisation par cette dernière de l'approvisionnement en gaz comme une arme de guerre. La flambée des prix du gaz qui en a découlé s'est répercutée sur le prix de l'électricité produite dans les centrales et, par ce biais, sur les prix de l'électricité en général. La corrélation entre le prix du gaz et le prix de l'électricité, due au principe de la préséance économique, ou,

S'il existe des raisons objectives de critiquer ce mécanisme de fixation du prix de l'électricité au niveau européen, c'est précisément parce que la question de la sécurité des approvisionnements énergétiques

au détriment d'une vision à plus long terme d'une meilleure indépendance énergétique de notre continent. Nous avons facilité la consommation au détriment des investissements dans la production d'électricité, car ceux-ci créent, évidemment, un coût final plus élevé.

On oublie cependant que nous en avons beaucoup bénéficié, à l'échelon national, jusqu'à la guerre en Ukraine et que le mécanisme de la préséance économique a aussi largement contribué au développement des énergies renouvelables. On oublie également que nombre des dysfonctionnements constatés aujourd'hui proviennent de la manière dont nous avons géré la libéralisation du secteur, essentiellement au profit des distributeurs d'électricité plutôt qu'au profit des producteurs. La loi Nome, adoptée par le Parlement français en 2010, est loin d'avoir rempli ses objectifs en matière de diversification de l'offre de production et a même entraîné certains effets spéculatifs, justement dénoncés par notre collègue Fabien Gay.

après l'invasion de la Crimée, à nous opposer à la construction du gazoduc Nord Stream 2, qui accroissait significativement notre dépendance énergétique à la Russie.

d'État chargée des affaires européennes, que nous avons auditionnée ce matin en commission des affaires européennes, nous l'a confirmé : cette réforme tendra à faire baisser les prix et à les rendre moins volatils sans sacrifier la transition énergétique, notamment en faisant en sorte que le principe de préséance économique

importé de l'électricité grâce à l'interconnexion des réseaux et à l'existence d'un marché de gros garantissant des prix corrects. Je vous invite, chers collègues, à étudier de près la situation énergétique du Royaume-Uni,

Indéniablement- tous nos compatriotes en vivent les difficultés, dans leur quotidien ou dans leurs entreprises -, le marché européen de l'électricité n'a pas répondu aux objectifs initiaux qui lui étaient assignés. Le principe de la concurrence libre et non faussée n'a pas diminué le prix de l'électricité. Il alimente l'inflation et n'a en rien permis de lutter contre la précarité énergétique. En France, il a même conduit à l'affaiblissement d'EDF, le plus important énergéticien d'Europe et l'un des premiers au monde. À dessein, ou faute de pilotage stratégique de la part l'État, actionnaire majoritaire, EDF a été sacrifiée sur l'autel de la concurrence. Ce qui fonctionnait jusque-là et participait grandement de notre souveraineté industrielle nationale a été déconstruit et affaibli. Je le rappelle, le critère d'évaluation de la réussite du développement du marché était non pas le prix ni la qualité du service, mais la quantité et la proportion de l'électricité vendue par des fournisseurs alternatifs à EDF. fournisseurs alternatifs n'ont jamais respecté l'obligation initiale qui leur était faite de produire par leurs propres moyens de l'électricité. Du négoce, du commerce

une envolée croissante des prix, alimentée par une crise de l'offre et des pratiques de spéculation qui ont largement enrichi les des marchés de l'énergie. Si certains consommateurs se sont appauvris et ont plongé dans la difficulté, d'autres acteurs en ont fait leur richesse.

Dans ce contexte extrêmement préoccupant, qu'attendons-nous du Gouvernement, non pour résoudre les difficultés de l'instant, auxquelles il apporte quelques solutions conjoncturelles, mais pour répondre aux problèmes structurels du marché de l'électricité ? C'est la question que soulève cette proposition de résolution, dont nous partageons totalement les constats. L'électricité L'électricité n'est pas un bien marchand comme un autre. Elle est d'abord, plus que tout autre produit, au coeur de la civilisation, et elle le sera plus encore avec le temps, eu égard aux transitions que doit opérer notre société pour être au rendez-vous climatique de la neutralité carbone en 2050. On la retrouve de l'alimentation aux transports, en passant par l'habitat. Elle est absolument partout, comme le sont depuis plus de deux siècles les énergies fossiles. Ne se stockant pas à grande échelle, elle nécessite un ajustement parfait et permanent entre la production et la consommation. En définitive, l'électricité est un bien commun,

Les prix doivent être indépendants du marché des énergies fossiles. La proposition de résolution invite à extraire le marché de l'électricité de la concurrence. Nous pensons que, si cette option doit être privilégiée, des régulations spécifiques doivent aussi être envisagées. chaque fois que nous interrogeons le Gouvernement sur ses propositions de réforme structurelle du marché, qu'il défend au sein des instances européennes, aucun début un tant soit peu concret de réponse ou d'orientation ne nous est apporté. Madame la ministre, prenez vos responsabilités pour défendre l'intérêt général des Français à Bruxelles,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà plus de quinze mois que la folle envolée des prix de l'énergie déstabilise le pouvoir d'achat des Européens et des Français, asphyxie les budgets de nos communes et menace la vie économique de nos entreprises. Et depuis quinze mois, économistes, experts ministres- à commencer par Bruno Le Maire, ici même, à plusieurs reprises -s'accordent sur un point : il y a un problème avec l'organisation actuelle du marché européen et la fixation des prix de l'électricité. Or, depuis quinze mois, rien ne se passe. Avec cette Avec cette proposition de résolution, nous vous proposons d'envoyer un signal fort pour dire : « Ça suffit ! La France ne veut plus du système actuel de fixation des prix. En réalité, le problème est structurel. La hausse a été forte et continue bien avant la guerre en Ukraine. La déstabilisation récente n'a fait que révéler des failles profondes, liées aux mécanismes de libéralisation et de privatisation, qui ont enfermé les marchés gazier et électrique dans des logiques concurrentielles court-termistes. du marché- -inventée par strates successives par les instances européennes a imposé une concurrence artificielle contraire à la rationalité économique du secteur de la production et de la distribution de l'énergie.

C'est pourquoi la sortie de ces mécanismes concurrentiels, sans rapport avec les réalités industrielles de la production, est urgente. Il est impératif non seulement de décorréler le prix de l'électricité de celui du gaz, mais aussi d'organiser la sortie de ces mécanismes pour revenir à une politique tarifaire

Cette sortie est d'autant plus indispensable qu'une stabilité retrouvée des prix, plus conforme à nos coûts de production, est indispensable. Il s'agit tant de garantir la souveraineté industrielle nécessaire à la sécurité de notre approvisionnement, que de planifier les investissements massifs supposés par la décarbonation. Sans vision de long terme, nous allons dans le mur. Or ce marché est organisé sur le court terme Nous ne pouvons plus accepter que ce bien universel essentiel soit confisqué par des logiques de profit aveugle. La volatilité des prix obère les investissements dans le système électrique, ainsi que ceux nécessaires à la transformation écologique. Elle dilapide les fonds publics dans des boucliers tarifaires, qui créent autant de trous qu'ils n'en bouchent, tout en continuant à financer des acteurs spéculatifs, alors que la garantie d'un prix stable réglementé offrirait à tous, particuliers, entreprises et collectivités locales, une meilleure sécurité. Nous proposons, vous le savez, de revenir à un monopole public capable d'évaluer les coûts marginaux à long terme de ses différentes unités de production, ayant la maîtrise de son programme d'appel.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier les auteurs de cette proposition de résolution, qui nous offrent l'occasion, après avoir débattu des tarifs réglementés pour les collectivités en décembre, d'aborder une nouvelle fois les problématiques du marché européen de l'énergie. Mon collègue Franck Montaugé a exprimé les nombreuses aberrations de ce marché, qui, bien loin de réaliser ses promesses de réduction des factures des consommateurs, n'aura servi qu'à la spéculation et à la multiplication de fournisseurs alternatifs. Il a également insisté sur la nécessité de considérer l'électricité comme un bien commun devant être décorrélé des logiques du marché. Madame la ministre, si vos promesses de restructuration d'EDF aboutissent, ne perdez pas de vue ce principe fondamental pour nos concitoyens et pour l'intérêt général. Les textes, nationaux la crise énergétique, passent les uns après les autres, mais ils ne sont que des rustines ne répondant aucunement aux tendances structurelles et aux graves dysfonctionnements du marché européen de l'énergie. Les mesures du Gouvernement restent profondément ancrées dans cette logique de marché et ne permettent que d'en combler les insuffisances par de l'argent public. Comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de résolution, la remise en cause d'une politique tarifaire décidée par l'État et l'abandon des coûts de production comme élément de la base de calcul des prix de l'électricité au profit d'un prix formé sur le marché expliquent l'impasse dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Pendant ce temps-là, les consommateurs finaux, particuliers et professionnels, continuent de subir l'explosion de leurs factures, qui se répercute directement sur leur budget du quotidien et sur leurs coûts de production. Je pense également aux collectivités territoriales, qui, depuis de nombreux mois, réalisent des efforts importants pour réduire leur consommation et ainsi tenter de préserver les budgets Ainsi, quand le marché devient obsolète, pour reprendre les mots de votre collègue Bruno Le Maire, et que les conséquences sont majeures pour nos concitoyens, il est du devoir du Gouvernement et des pouvoirs publics de réfléchir immédiatement à la refonte ou à la sortie de ce système.

les récents exemples de l'Espagne et du Portugal, qui ont eu l'autorisation de déroger aux règles européennes pour fixer les prix de l'énergie en fonction de leur propre mix énergétique, sont particulièrement intéressants. Cela a fait baisser les factures d'électricité des Espagnols et des Portugais de 10 % à 20 %. La spécificité géographique de ces pays justifie certainement ces adaptations, mais cette dérogation temporaire prouve que ce sont le marché et les interconnexions qui tirent les prix vers le haut. Alors que notre mix énergétique se base très largement sur nos capacités nucléaires et sur les énergies renouvelables, que nous espérons voir se multiplier dans les années à venir, il est de notre intérêt de demander une dérogation similaire pour tirer profit de nos choix énergétiques.

activement les négociations européennes sur le marché de l'énergie. Il est particulièrement dommage que la présidence française du Conseil de l'Union européenne n'ait pas permis d'avancer sur le sujet. Même si certains points de cette résolution mériteraient d'être un peu nuancés, notamment pour permettre des négociations avec nos partenaires européens, nous approuvons pleinement l'objectif de sortie du système électrique des mécanismes concurrentiels. La parole

Il me semble indispensable de la lire au regard du contexte dans lequel nous nous trouvons et de ses implications sur le système électrique français. Le contexte immédiat, c'est tout d'abord celui d'une crise climatique et d'une crise énergétique sans précédent depuis plus de quarante Cette crise sur la sécurité d'approvisionnement m'a conduite à prendre des mesures exceptionnelles pour passer l'hiver dans les meilleures conditions- plan de sobriété, sécurisation de nos importations et de nos interconnexions et augmentation des marges de manoeuvre sur les moyens de production d'électricité existants -notamment votées par votre assemblée cet été. Je rappelle que la sécurisation de nos importations est aussi liée au bon fonctionnement du marché européen de l'électricité. Lorsqu'on prétend en sortir, on pose la question de ce bon fonctionnement.

au moment où les consommateurs anticipaient des ruptures d'approvisionnement, intégrant cette prime de risque dans les coûts. C'est très grave ! Nous connaissons tous les effets de ces hausses historiques pour les Français, les entreprises et les collectivités locales. C'est pourquoi le Gouvernement a pris un engagement très clair : nous ne laisserons tomber personne ! C'est aussi la raison pour laquelle nous avons pris des mesures exceptionnelles pour protéger le pouvoir d'achat des Français et la compétitivité de notre économie

C'est bien la raison pour laquelle je défends, face à mes homologues européens, une position forte au nom de la France : celle d'une refonte équilibrée du marché européen de l'électricité. Cependant, je veux être claire nous ne souhaitons pas sortir du marché européen de l'électricité. Ne cédons pas aux fausses bonnes idées, car ce sont toujours les plus nocives pour notre pays. Ainsi, nous devons préserver les avantages actuels du marché, dans l'intérêt des consommateurs et de la lutte contre le réchauffement climatique.

La Commission européenne a annoncé qu'elle travaillait désormais en ce sens. Une proposition législative européenne est attendue pour le premier semestre 2023, à l'occasion du conseil des ministres de l'énergie.

aux deux tiers d'énergies fossiles qui ne sont pas présentes sur notre territoire, il faut accepter une logique de marché, l'alternative étant une logique de pénurie. Dans ce cadre, nous devons maximiser cette production décarbonée avec une meilleure organisation de marché, de marché, concurrentielle ou plus régulée en fonction des spécificités des technologies. Pour les nouvelles énergies renouvelables, la concurrence baisse les coûts de production et met les porteurs de projets au défi de produire au coût le plus bas,

et de la spécificité du parc nucléaire français, ainsi que du fait qu'il n'y a qu'une technologie de réacteur de forte puissance en Europe. Je tiens ici à saluer tous les salariés de la filière : ce sont leurs efforts, conjugués à ceux de tous les Français dans la sobriété énergétique, qui nous permettent de réussir le passage de l'hiver.

sont une reconnaissance du fait que l'électricité est un bien de première nécessité pour les ménages et les très petites entreprises. Ils constituent une offre universelle, dont peuvent bénéficier tous les consommateurs, sans condition de ressources ou de solvabilité. Ils sont enfin une référence tarifaire

aux ménages et aux très petites entreprises au prix le plus bas d'Europe. Protéger le consommateur, c'est s'assurer que son fournisseur, quel qu'il soit, prenne ses responsabilités. C'est s'assurer qu'il se couvre quand il s'engage sur le long terme, qu'il prend des engagements de production, qu'il participe au déploiement du mix décarboné dont nous aurons besoin demain. c'est s'assurer que les fournisseurs anticipent les défis des dix prochaines années, de sorte que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Mais c'est aussi leur garantir des prix qui couvrent les coûts complets de notre système énergétique, sans marges excessives ni rentes de situation. on peut se demander si la future régulation ne devrait pas fixer un cadre minimum à la politique de couverture, afin que cette dernière repose davantage sur des signaux-prix prévisibles à long terme.

tenus de prendre leur part dans leur production et dans les charges de service public. Là où le gouvernement en place en 2010 avait fixé des obligations fortes à EDF sans véritablement les contrebalancer par de nouveaux devoirs pour ses concurrents, nous équilibrerions ces droits et ces devoirs. Ces quelques éléments me semblent montrer sans aucune ambiguïté qu'une réponse sur le principe de la concurrence dans notre système électrique ne peut pas être simpliste, au risque d'être grossièrement inexacte. Elle me semblerait tout aussi imparfaite qu'une doxa idéologique qui revendiquerait la concurrence pour la concurrence. La question porte non pas tant bien-fondé de la concurrence, mais sur la création d'un cadre de marché dans lequel le jeu de la concurrence permettrait d'atteindre nos objectifs communs de politique publique de long terme, au meilleur coût pour la collectivité et pour les citoyens. C'est bien la feuille de route que je me suis fixée à la tête de ce ministère. C'est la position que je défendrai dans les discussions du texte que proposera la Commission européenne au premier semestre de 2023. Pour toutes ces raisons, je vous invite à ne pas voter cette proposition

du groupe Les Républicains. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

vert » ; Projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (procédure accélérée